d'atténuation » et transitoire sur 2019 et 2020, nous proposons purement et simplement de revenir au régime pérenne dont bénéficiait jusqu'ici le secteur agricole, notamment l'arboriculture, le maraîchage ou encore la viticulture, qui emploient massivement des travailleurs saisonniers. Il serait Il serait facile de reprendre les termes de notre cher ministre de l'agriculture, qui critiquait en septembre dernier, sur ces mêmes travées, cette « mesure technocratique et mortifère » lors d'une question d'actualité au Gouvernement

et ce même si l'Assemblée nationale a décidé de réintroduire l'exonération jusqu'à 1,15 SMIC avec un point de sortie à 1,6 SMIC. Comment, en effet, régler le problème de l'important recours aux heures supplémentaires ? Nous savons tous qu'en raison de la courte saisonnalité de ces produits les semaines sont très chargées et dépassent allègrement les trente-cinq heures légales. Il est tout de même étonnant de constater que le Gouvernement souhaite ici saper une mesure favorable à la compétitivité de nos agriculteurs. Nous souhaitons donc maintenir le dispositif TO-DE dans son régime actuel et de façon pérenne, pour permettre à nos agriculteurs de faire face à la concurrence internationale et au. Le système a fait la preuve de son efficacité pour lutter contre le travail clandestin. En restant sur vos positions, monsieur le ministre, vous risquez de fragiliser, voire de mettre en péril nombre d'exploitations agricoles qui n'ont vraiment pas besoin de cela. C'est aussi prendre le risque d'accroître, ici et là, le malaise agricole en remettant en question l'un des piliers de l'emploi dans nos territoires ruraux. Pour 40 millions d'euros, qui, rapportés au budget total du projet de loi de financement de la sécurité sociale, semblent bien dérisoires, le Gouvernement s'accroche et ne veut pas concéder son erreur, au mépris des réalités profondes et complexes du travail et du secteur agricoles. durable et accessible à tous, c'est un nouveau signal négatif que vous envoyez à nos agriculteurs. C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir voter le retour au dispositif actuel d'exonération pour les travailleurs saisonniers.

occasionnels et de demandeurs d'emploi pour les entreprises réalisant des travaux agricoles en tant que prestataires extérieurs. Les entreprises de travaux agricoles sont exclues de ce dispositif depuis 2015 et cette perte n'a jamais été atténuée par le recours au dispositif « bas salaire »- malgré les projections du gouvernement de l'époque. Ces entreprises ne comprennent pas pourquoi l'exonération ne s'appliquerait pas aux travaux agricoles qu'elles réalisent pour le compte des exploitants agricoles.

Sur certains territoires, c'est le cas du mien, les entreprises de travaux agricoles se développent. Elles participent de la stratégie de certaines exploitations. C'est une forme de mutualisation sur certains territoires et pour certains types de travaux. Leur coût, évidemment, est répercuté dans celui des exploitations qui font

à la même enseigne : entreprises agricoles et entreprises de prestations agricoles. La situation actuelle de ces dernières est particulièrement injuste : elles réalisent des travaux semblables, ont recours bien souvent au même type de main-d'oeuvre, mais elles ne sont pas éligibles au même dispositif. En 2015, le Gouvernement sortait ces entreprises du dispositif conçu pour les TO-DE en avançant des projections qui se sont révélées erronées, le raisonnement étant que le dispositif « bas salaires »- la réduction « Fillon » -allait prendre le relais et compenser. Cela n'a pas été le cas. Je propose donc que nous soyons cohérents en adoptant cet amendement. Les

vise à supprimer les différents alinéas qui correspondent à la dégressivité et à la suppression, à terme, après 2021, du

Il fallait changer de modèle, faire plus de bio, utiliser moins de produits phytosanitaires et moins de pesticides, supprimer le glyphosate, etc. Monsieur le ministre, c'est totalement contradictoire ! Supprimer le TO-DE aujourd'hui ou le faire

À cet égard, je rappelle que tous nos amendements, du coefficient multiplicateur à la mise en place d'indices publics de construction du prix ou encore de prix plancher par production, ont été rejetés.

Aussi, faute d'actions d'envergure concrètes et pérennes, nous en arrivons à des mesures de sauvetage comme celles qui sont proposées aujourd'hui. C'est pourquoi je défends cet amendement, comme d'autres dans l'hémicycle, qui vise à préserver de manière exceptionnelle les allégements de cotisations spécifiques dont sont bénéficiaires actuellement les exploitants agricoles employant de la main-d'oeuvre saisonnière. Nous le savons, dans un certain nombre de productions agricoles, le recours à la main-d'oeuvre saisonnière est une nécessité

C'est pourquoi, pour l'heure, nous proposons de maintenir ce dispositif, en attendant des mesures équivalentes plus acceptables et un véritable statut du travailleur saisonnier, afin de ne pas favoriser le retour à une pratique trop largement répandue, dans ce secteur comme dans d'autres,

L'article 8 du projet de loi supprime ce dispositif TO-DE au motif qu'il serait moins attractif que l'allégement général de charges envisagé avec la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le Conscient de la difficulté que poserait cette suppression pour certaines exploitations, le Gouvernement a fait adopter un amendement visant à atténuer les effets de la suppression du dispositif TO-DE au titre des années 2019 et 2020. En l'état actuel, la mesure d'atténuation proposée ne compense pas intégralement la suppression du CICE et du dispositif TO-DE.

le seuil de dégressivité prévu à l'article 8, pour le porter à 25 % pour 2019 et 2020. Une telle modification laisserait deux ans aux différentes parties prenantes pour trouver une solution pérenne.

subir. Ainsi, l'exonération des rémunérations versées aux travailleurs saisonniers serait totale jusqu'à une rémunération de 1,25 SMIC en 2019 et en 2020, tout comme dans le régime actuel.

Ces exonérations sont cruciales pour les filières agricoles- arboricole, viticole, maraîchère et horticole. Elles leur permettent de conserver de la compétitivité face à des pays aux coûts salariaux plus faibles. Le Gouvernement veut supprimer le TO-DE en le remplaçant par un renforcement immédiat de l'allégement général des charges, mais force est de constater que le compte n'y est pas encore, et ce malgré les avancées obtenues lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, où a été prévu un plateau d'exonération à 1,15 En effet, le dispositif actuel ne permet pas de compenser suffisamment le basculement des exonérations spécifiques. Avec mes collègues du groupe du RDSE, après nous être pleinement mobilisés pour le maintien du TO-DE,

: comme je l'ai dit en introduction, ces exonérations apportent de la compétitivité aux filières les plus exposées. Je suis d'ailleurs un peu inquiet : tels que les débats se profilent, je crains que les amendements adoptés ici ne soient rejetés par l'Assemblée nationale. Notre amendement permet de concilier les intérêts de la filière agricole avec les objectifs du Gouvernement en prolongeant les avancées obtenues lors du débat à l'Assemblée nationale.

La défense de tous ses amendements et l'émoi qu'a suscité la proposition du Gouvernement montrent à quel point il était important

exonérer, c'est décider une perte de recettes pour la sécurité sociale. Nous avons toujours essayé de maintenir cet équilibre en commission, et nous vous demandons de réfléchir à ces deux aspects qui est propre à la profession agricole, que nous ne mésestimons pas ; et celui de l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. J'avais d'ailleurs proposé

c'est-à-dire une exonération totale à 1,25 SMIC si nécessaire- et ça me paraît l'être -pour des filières comme les fruits et légumes et la viticulture.

Aujourd'hui, le Gouvernement n'entend pas revenir sur le TO-DE dans son ensemble, puisque la volonté est de baisser les charges. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a accepté un « tampon », qui assure une

inquiets de constater que, face à une situation économique et sociale difficile pour bon nombre de territoires et dans maints secteurs, les propositions se sont multipliées pour priver notre système de sécurité sociale de cotisations versées par les entreprises, toujours dans un souci affiché de préserver l'emploi, monsieur le ministre. Vous devez tout de même être satisfait, car la petite musique que vous jouez depuis votre prise de fonctions, même si vous n'êtes pas ministre depuis longtemps, s'insinue dans les esprits. petite musique reprend les mêmes partitions que vos prédécesseurs : il faut diminuer le coût du travail et fiscaliser la sécurité sociale, et il est hors de question de chercher des recettes nouvelles. Toutes nos propositions sont rejetées, qui pourtant tendraient à redresser la barre, même quand il s'agit de faire respecter la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Alors, allons-y, ouvrons la boîte de Pandore, et que chacun et chacune formulent des propositions d'allégements de cotisations sociales Qu'en est-il de la situation spécifique des travailleurs saisonniers ? Le travail saisonnier, sur lequel mes anciens collègues Annie David et Dominique Watrin s'étaient investis, connaît effectivement des problèmes particuliers. Je souscris à ce que mes collègues ont dit à son sujet : la grande précarité des travailleuses et des travailleurs saisonniers nécessite de prendre des mesures positives, comme le versement de la prime de précarité, la reconduction des contrats pour les salariés volontaires, le droit au logement, l'accès à la formation et l'augmentation des moyens donnés à l'inspection du travail pour lutter contre le travail non déclaré- Cécile Cukierman en a parlé. Sur ce dernier point, je veux rappeler que, malgré les exonérations de cotisations, le travail non déclaré est extrêmement répandu chez les saisonniers agricoles. Pour certains gros agriculteurs qui ne recherchent que la productivité et la flexibilité de la main-d'oeuvre, la concurrence entre les travailleuses et les travailleurs est un moyen de pression des salaires et des droits sociaux Ce n'est pas en réduisant les moyens de l'inspection du travail que les choses s'amélioreront. Or, par exemple, plus d'une vingtaine de postes d'agents contrôleurs ont été supprimés dans la région Grand Est en 2018. Cette situation est complexe et dramatique. Nous ne pouvons rester sans rien faire dans l'immédiat, compte tenu des choix, essentiellement politiques, que

La main-d'oeuvre saisonnière représente environ 70 % de l'ensemble des salariés agricoles et 22 % de volume du travail. Le secteur viticole est sans conteste le premier employeur de travailleurs saisonniers. En 2016, la masse salariale des 452 283 contrats TO-DE signés s'élevait à plus de 600 millions d'euros.

Je rappelle que, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, un dispositif compensant partiellement la suppression du TO-DE a été adopté, permettant une exonération des cotisations patronales- totale jusqu'à 1,15 SMIC, puis dégressive jusqu'à 1,10 SMIC -pour les années 2019 et 2020. C'est une avancée, mais celle-ci ne suffira pas à compenser intégralement le coût supplémentaire induit par la suppression du TO-DE et la fin du CICE. De plus, ce dispositif n'est que transitoire. Les pertes sont estimées à 39 millions d'euros pour l'ensemble de l'agriculture et à 12,8 millions d'euros pour la viticulture en cas d'application du dispositif proposé par l'Assemblée nationale.

des emplois saisonniers. Hier, j'ai pris l'exemple des pépiniéristes viticoles. Ils sont 600. À la force des bras, ils sont devenus l'année dernière mondiaux.

embauchent, emploient nos concitoyens et font parfois survivre des familles de nos communes. Nous leur devons ce combat.

qui vous donne rendez-vous lors de l'examen du projet de loi de finances pour trouver les millions d'euros manquants, me semble particulièrement intéressante. Monsieur le ministre, montrez-nous que votre plaidoyer pour l'agriculture

Monsieur le ministre, je vous ai entendu. Je sais l'intérêt que vous portez au milieu rural et à l'agriculture. J'ai pour vous beaucoup de respect et d'estime. Vous avez été, comme un certain nombre d'entre nous, président de département, donc tout près de la ruralité.

L'économie agricole du département de l'Aisne se développe surtout sur de grandes plaines céréalières et betteravières. Mais elle comporte, dans les vallées et dans certains secteurs, une activité de viticulture, avec la production de 10 % du champagne français, ainsi que différentes activités maraîchères : légumes, fruits, aromates, safran bio ... Ces

la fin de l'exonération va créer des problèmes majeurs et déstabiliser des filières entières. Monsieur le ministre, le 26 septembre dernier, ici même, nous avons tous applaudi sincèrement vos propos lorsque vous avez, en tant que sénateur, interpellé le ministre.

ministre est et sera un très bon ministre de l'agriculture, parce qu'il est imprégné d'agriculture. Son département, qui est

par le maraîchage et la culture biologique, les vergers de l'Orléanais, l'arboriculture, la vigne, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces activités seront fortement touchées si le Gouvernement va au bout de son raisonnement. Je voulais simplement le signaler,

dans les départements les plus concernés- mais je crois que nous sommes tous concernés, peu ou prou, par les cultures maraîchères, par les fruits et les légumes.

Le scrutin est clos.

où nous avons consacré le principe du bulletin de paie unique. Qu'est-ce qu'un bulletin de paie unique ? Il s'agit pour l'employeur de n'émettre qu'un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, mais à cheval sur deux mois distincts.

En 2017, quelque 54 % de la presse quotidienne régionale et 13 % de la presse quotidienne nationale recourent au portage pour la distribution des titres, soit 800 millions d'exemplaires par an. Le portage emploie 12 000 porteurs. Il représente un enjeu crucial pour le débat démocratique, pour la presse, notamment locale, et pour la diffusion de l'information dans l'ensemble des territoires. Comme tous les secteurs économiques, le portage a bénéficié du CICE, qui lui a permis de recruter et d'investir dans des outils d'amélioration des performances. Or, en l'état actuel, la transformation du CICE en allégements de charges ne pourra pas bénéficier aux entreprises de portage de presse,

qui causerait de très forts risques pour l'équilibre économique du portage. La volonté du législateur étant de compenser intégralement la suppression du CICE, il serait incohérent que les entreprises de portage soient privées d'une telle compensation. Il convient donc de préciser la portée de l'interdiction

En outre, depuis 2009, les employeurs sont exonérés de cotisations patronales sur les rémunérations versées aux vendeurs, colporteurs et porteurs de presse. L'exonération est applicable aussi bien sur l'assiette forfaitaire que lorsque les cotisations sont calculées sur le montant des rémunérations réelles. Ainsi, le cumul de ces dispositifs aboutit à un coût du travail extrêmement faible. Permettre le cumul de ces dispositifs avec les allégements généraux reviendrait à accorder auxdits employeurs un avantage exorbitant. C'est pour éviter ces situations que le cumul

à prestations définies, versées notamment aux cadres dirigeants de plusieurs entreprises importantes. Je nous invite collectivement à ouvrir les pages de ce que l'on appelle un « document de référence », c'est-à-dire le document de promotion que les grands groupes inscrits à la cote officielle de la bourse mettent en circulation pour narrer le roman de leur entreprise. Regardons de près le document de Danone, celui d'Engie ou de n'importe quelle autre entreprise un chapitre y est toujours consacré à la gouvernance, notamment au dispositif mis en place pour fidéliser les administrateurs de ce type d'entreprise. Nul doute qu'entre les plans d'achat, les plans d'action de performance, les jetons de présence, les éléments de rémunération variable, les plans de retraite à prestations définies et les rémunérations annuelles à

Emmanuel Faber, dont la retraite sera calculée sur la base de plus de 2 millions d'euros. Voilà qui est assez éloigné, nous en conviendrons toutes et tous, de ce qui est pratiqué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

il ne convient pas de basculer au-delà de la taxation cumulée, qui est considérée comme confiscatoire par le Conseil constitutionnel. Je précise, par ailleurs, qu'il s'agit de contributions spécifiques s'appliquant à des personnes

vous proposez d'augmenter à hauteur de 34 % le taux de contribution. Nous rappelons que le Conseil constitutionnel avait déjà censuré une contribution établie à 21 % pour la part des rentes supérieure à 24 000 euros par mois. En effet, le cumul entre l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et la contribution salariale spécifique au taux de 21 % pour la fraction des retraites chapeau excédant 24 000 euros, aboutissait à un taux d'imposition de 75 %, jugé confiscatoire par le Conseil. Au regard de cette jurisprudence, nous sommes défavorables

encore ce matin en commission des affaires économiques. Mais si, mes chers collègues, il y a de l'argent, et même beaucoup, dans ce pays, mais il est accaparé par une minorité ! Et cette réalité est de plus en plus criante

L'association entre un médecin retraité et un médecin en activité ou un médecin en recherche d'installation en est une. Elle permet d'apporter une réponse au problème de la transmission et d'avoir une prise en charge continue entre un médecin et son successeur sur des territoires fragiles en termes de couverture. Pour cela, l'amendement vise à mettre en place une exonération fiscale à hauteur de 50 000 euros nets annuels pour le médecin retraité.

Je les voterai, car, à l'heure actuelle, l'incitation est insuffisante. Bien que cela soit difficile à évaluer, il y a probablement un gisement de temps médical mal exploité.

activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite [ ...] ». Or je n'ai pas le souvenir qu'un chiffre d'affaires soit soumis à cotisations sociales. Il s'agit donc de revenus. Et lorsque l'on parle de 90 000 euros de revenus, cela correspond à 7 500 euros par mois en plus de la retraite.

Nous avons décidé de faire évoluer ce plan en fonction des remontées du terrain des trois délégués, qui viennent de nous présenter leur rapport. Nous sommes en train d'instruire leurs recommandations, évidemment sur le cumul emploi-retraite, mais aussi sur ces trente ou quarante autres mesures du plan d'accès aux soins. Nous avons considéré que c'était dans le cadre de ce comité de suivi, avec l'ensemble des parties prenantes, prendrions les décisions quant à l'évolution des dispositifs visant à faciliter l'accès à du temps médical sur les territoires. Je trouve quelque peu bizarre que la Haute Assemblée se saisisse d'une seule mesure,

un rapport tous les six mois. J'estime que ce n'est pas le bon endroit pour discuter de l'amélioration de l'accès aux soins. Nous avons mis en place un comité de suivi très robuste, qui s'est engagé à faire évoluer les mesures. Il me semble plus légitime que les professionnels eux-mêmes, les parties prenantes elles-mêmes, s'emparent des mesures qu'il semble important de mettre en oeuvre. Le Gouvernement s'est engagé à suivre les recommandations du comité de suivi, et nous le faisons. Là, je m'engage à travailler sur le cumul emploi-retraite pour le faire évoluer.

l'exemple d'un médecin retraité qui se rend compte des problèmes auxquels sont confrontées tant sa profession que les zones rurales, et décide de reprendre du collier. Soit dit en passant,

réduction générale de cotisations patronales étendant le dispositif Fillon aux contributions de retraite complémentaire dès le 1 janvier 2019 et aux cotisations d'assurance chômage à compter du 1 octobre 2019. Actuellement, les cotisations patronales d'assurance maladie s'élèvent à 13 demain, c'est-à-dire en 2019, les employeurs bénéficieront d'un taux réduit de 7 %. Avec l'annonce de la suppression des cotisations patronales au niveau du SMIC, il y a un véritable danger de voir les cotisations patronales disparaître totalement du financement de la sécurité

patronales, qu'est-ce qui justifie la présence des organisations professionnelles d'employeurs au sein des conseils de la sécurité sociale- soyez logiques ! -et, en premier lieu, du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ? D'un côté, le patronat demande la suppression des « charges sociales » et, de l'autre, il continue de codiriger les caisses de la sécurité sociale, alors même qu'il y participe

Ce que vous faites aujourd'hui en supprimant totalement les cotisations patronales sera non seulement inefficace pour la création d'emplois, mais surtout très dangereux pour le maintien du paritarisme. C'est la raison pour laquelle nous défendrons plus loin, à l'article 19, un amendement visant à rétablir les élections des caisses de la sécurité sociale.

Mme Jocelyne Guidez. Comme les entreprises ultramarines qui cumulent différents soutiens à l'emploi tels que la transformation du CICE en allégement de charges, le particulier employeur bénéficie actuellement d'un dispositif fiscal lui permettant de réduire le coût de l'emploi à son domicile, mais aussi d'allégements de charges sociales. Parmi ces dernières figurent celles qui sont prévues à l'article L. 735-3-2 du code de la sécurité sociale que le PLFSS pour 2019 entend supprimer. Cette suppression entraîne une augmentation du coût de l'emploi d'un salarié à domicile de 11 % pour les 60 000 particuliers employeurs. Elle risque de conduire à une augmentation drastique du travail non déclaré et à des suppressions d'emploi. Ainsi, cet amendement prévoit de porter la déduction de charges par heure déclarée de 3,70 euros aujourd'hui à 6,20 euros. Cette hausse significative a notamment pour objectif de rééquilibrer le coût de l'emploi à la suite de cette suppression d'allégements de charges prévues à l'article L. 735-3-2. De plus, ces employeurs ultramarins disposeraient de cette incitation pour recourir au dispositif du CESU et ainsi déclarer leurs salariés au réel. Cette mesure offre notamment l'occasion d'exprimer la confiance à l'égard des employeurs et de leur capacité à créer de l'emploi. Quel est l'avis de la commission ? Madame

à Mme Laurence Cohen. L'orientation politique du Gouvernement en matière d'emploi, comme celle d'ailleurs des gouvernements antérieurs, se polarise sur le coût du travail. Je l'ai déjà dit : pour nous, le travail n'est pas un coût. Quand on procède à l'allégement des cotisations sociales, c'est la rémunération du travail elle-même qui baisse- faut-il le rappeler ici ? Par voie de conséquence, la contribution apportée par le travail au financement de la sécurité sociale constitue une amélioration du pouvoir d'achat. Les exonérations de cotisations sociales patronales mettent en péril le financement durable de la sécurité sociale, faisant de nos lois de financement des parcours d'austérité permanente. L'équilibre ne se finance que par la réduction des droits et ouvre en grand toutes les « trappes à bas salaires » qui engloutissent chaque année un peu plus les salariés, les femmes d'abord- je l'ai déjà dit dans cet hémicycle -, les aspirations des plus jeunes, le respect de leur formation et bien d'autres choses. Il faut donc réduire la part des exonérations accordées aux entreprises qui font des bas salaires, en quelque sorte, leur viatique et l'essence de leur politique de rémunération. Quel est l'avis de la commission

En 2007, a été mis en place un système d'exonération des cotisations employeurs pour les associations et les organismes d'intérêt général, notamment dans les zones de revitalisation rurale.

suite de l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale. Cet article exclut de l'assiette du forfait social les indemnités de rupture du contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective ou d'un congé de mobilité. Je le rappelle, le forfait social est une contribution à la charge de l'employeur, qui a été instaurée initialement afin de réduire le déficit de la sécurité sociale, suite d'une recommandation de la Cour des comptes. Puisque tout ce projet de financement de la sécurité sociale est fondé sur l'idée de désendettement, il nous paraît peu opportun de supprimer cette contribution. Alors que les prestations sociales ne sont que peu revalorisées, alors que la hausse de la CSG pour les retraités est maintenue, alors qu'un certain nombre d'aides pour les personnes en situation de handicap ont été supprimées, les entreprises, elles, bénéficient de cadeaux fiscaux. Au titre de l'année 2018, elles reçoivent 20 milliards d'euros de crédit d'impôt compétitivité et emploi. En 2019, la transformation du CICE en allégements de cotisations leur permettra d'économiser là encore 20 milliards d'euros. Les entreprises n'ont pas besoin d'allégements supplémentaires de leurs charges. Le Gouvernement demande aux plus précaires de mettre la main à la poche et de participer aux restrictions afin de permettre le désendettement de la sécurité sociale. Il nous paraît normal que les entreprises fassent de même et continuent de participer au désendettement de la sécurité sociale. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 8 et le maintien du forfait social. Quel

la nouvelle manière dont on pourrait imaginer le lien entre le capital et le travail, une vieille idée gaulliste mais pas seulement. Nous avons un désaccord de fond et vous ne serez pas vexée si je donne un avis défavorable à votre amendement, qui vise à supprimer la disposition en tant que telle pour ne plus jamais la revoir.

Il me semble dommage de renoncer à cette compétence législative. Par ailleurs, l'adoption de l'amendement du Gouvernement visant à l'alignement progressif en six ans

Que l'on se garde de me faire ce mauvais coup ! Comme l'écrivait Maupassant, le regard moderne sait voir la gamme infinie des nuances. Oh là là ! La France a protégé sa production viticole, son vin,

d'augmenter très vite les taxes pour éviter l'alcoolisation foetale, les violences faites aux femmes, les violences routières, les cirrhoses, les cancers

Il manque 2 000 hectares, madame, à mon seul pays. Il manque 2 000 hectares en Martinique : le rhum est exporté à 80 % dans une centaine de pays et seuls 8 % sont consommés par la population locale. Et on veut me faire croire que, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Atlantique, tous les Martiniquais sont couchés sous des cocotiers, boivent du rhum toute la journée- plus que les Français ne boivent de vin ! -et que nous sommes victimes de toutes les pathologies et de toutes les dérives comportementales liées à l'alcoolisation.

dans les DOM qu'en métropole. La réalité, c'est que l'Agence nationale de santé publique constate les dégâts en termes de santé sur la population.

particulièrement bien conçue présente dans les médias et sur internet et s'appuyant sur les professionnels de santé. À l'Assemblée nationale, le Gouvernement a amendé, nous en reparlerons dans le cours de la discussion, l'article 38

Cette affaire a été introduite à l'Assemblée nationale par un amendement quelque peu tardif et, là encore- c'est décidément la marque de votre gouvernement -, sans concertation.

pas à excuser une consommation frénétique d'alcool, mais on consomme moins d'alcools forts, et en particulier moins de rhum, en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion

Merci de conclure, chère collègue.

des addictions alcooliques qu'implique leur production. Pour cette raison, ils se sont unanimement- tout du moins ceux qui m'ont contacté -prononcés pour une contribution au financement des mesures de prise en charge des effets pervers de l'alcool dans le rhum. si la fiscalité pouvait, à elle seule, prévenir toutes les formes de consommation excessive, nous n'aurions pas ce débat, même s'il est certain qu'un prix trop accessible ne contribue pas à les enrayer. En d'autres termes, si les taxes permettaient de lutter contre l'alcoolisme ou le tabagisme, cela se saurait.

Partant de ce constat, la motivation de santé publique justifie que le surplus de la taxe soit affecté à un fonds dédié au financement de la prévention de l'alcoolisme et de la prise en charge de ses conséquences outre-mer. La place stratégique du rhum dans les économies ultramarines n'est plus à exposer. C'est dans cet esprit que j'évoquais l'idée d'un équilibre, ce qui nous amène à la problématique de l'étalement du surplus de la fiscalité. Un échelonnement sur dix ans permettrait en effet à la production de contribuer dès 2020, tout en bénéficiant d'un temps d'adaptation suffisamment long pour ajuster son modèle économique qui n'avait sans doute pas intégré la suppression d'une différenciation fiscale visant notamment à garantir un avantage comparatif au rhum.

La suppression de l'alignement progressif de la fiscalité sur les alcools forts dans les outre-mer sur celle qui est en vigueur dans l'Hexagone ne tient pas compte des enjeux de santé publique posés par la consommation de tels produits dans ces territoires, laquelle entraîne

texte par le rapporteur général en commission des affaires sociales prévoit un alignement que nous jugeons trop rapide, sans concertation avec les producteurs, et sans préavis. Pour rappel, les quatre territoires concernés ne regroupent pas moins de 23 distilleries. Au total, ce sont près de 15 000 emplois, directs et indirects, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui en dépendent. Compte tenu du marasme économique et du taux de chômage deux fois plus élevé dans ces territoires que dans l'Hexagone, il est indispensable de protéger cette filière et d'en sécuriser les emplois.

Le présent amendement a pour objet d'allonger le délai prévu dans l'article tel qu'il est proposé par le rapporteur général pour l'alignement de cette fiscalité afin de préserver l'équilibre entre les enjeux économiques et les enjeux de santé publique.

autrement dit par ceux qui connaissent le mieux leur territoire. Or ils se font battre par des gens qui parfois n'y ont jamais mis le moindre orteil. Nous serions donc non pas des citoyens à part entière, mais des citoyens entièrement à part. J'en prends acte.

l'alignement de la cotisation de sécurité sociale pesant sur les boissons alcooliques produites et consommées dans les départements d'outre-mer. Il tend à adapter le calendrier de convergence de la cotisation sur celle qui est applicable en métropole, en tenant compte compte à la fois des objectifs de santé publique et des nécessités d'adaptation du secteur de production.

outre-mer sur les alcools forts sur celle qui en vigueur dans l'Hexagone. Il uniformise aussi le mode de calcul de cette contribution de sécurité sociale en l'appliquant à un volume d'alcool pur

entre 2006 et 2013, selon les données de santé publique, ce que peut nous confirmer Mme la ministre. La préoccupation sanitaire est donc la même partout.

On connaît tous les bonbons Pina Colada ou Mojito et les autres substances alimentaires qui contiennent une référence à un produit alcoolique.

l'ensemble des produits dont la composition n'indique pas de produit mentionné à l'article 401 mais dont l'étiquetage des unités de conditionnement ou l'emballage extérieur comprennent des éléments ou dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit mentionné au même article 401.

Pour l'application des dispositions du présent code, sont dénommés produits alimentaires à référence alcoolique l'ensemble des produits dont la composition n'indique pas de produit mentionné à l'article 401 mais dont l'étiquetage des unités de conditionnement ou l'emballage extérieur comprennent des éléments ou dispositifs

sont celles qui sont les premières sanctionnées et les moins sensibles aux arguments présentés. Elle peut également s'adresser aux industriels,

: elle a raison, taxer n'a jamais changé le cours des choses

par un packaging festif, coloré et racoleur, particulièrement à l'égard des jeunes. Le propriétaire de la marque Rosé Sucette a notamment précisé : « Ces bouteilles, à moins de 3 euros sur linéaire, seront un tremplin permettant aux néophytes d'accéder aux vins plus classiques, notamment pour un public plutôt jeune et féminin ». À ce titre, les pouvoirs publics se sont intéressés à ce problème de santé publique dès la loi de finances pour 1997, en taxant ces boissons. Les chiffres de l'office français des drogues et des toxicomanies témoignent de l'efficacité de cette désincitation fiscale : en 1997, les ventes tombent à 100 000 litres contre 950 000 en 1996. Ce dispositif de politique fiscale a été renforcé en 2004 et a entraîné en 2005 une baisse de 40 % des ventes de prémix. C'est ainsi que les trois leaders du marché- Boomerang, Smirnoff Ice et Eristoff

Mais ces industriels se sont adaptés, en exploitant une faille de la loi de 2004 renforçant ce dispositif. En effet, cette dernière excluait du champ d'application de la taxe les vins aromatisés. Ainsi, des vins-coca ou des cidres aromatisés sont apparus sur le marché, ces derniers étant clairement adressés à la consommation des jeunes en raison notamment de leur marketing et de la politique de prix bas. C'est pour ces raisons de santé publique que le présent amendement prévoit d'étendre la taxe dite prémix aux boissons aromatisées à base de vin.

dans le même esprit que les deux précédents, vise à dénoncer les pratiques d'industriels qui cherchent à banaliser la consommation d'alcool par les jeunes. Les noms évocateurs de Rosé Sucette, Rouge Cola ou Bonbon Mojito prêtent à confusion et laissent croire que ces boissons sont anodines, ce qui est parfaitement irresponsable et inacceptable.

Une éventuelle modification du périmètre de cette taxe me semble devoir être précédée d'un travail en profondeur sur tous les paramètres. Comme je l'ai indiqué à l'Assemblée nationale, je suis d'accord pour travailler sur ces dispositifs et les améliorer,

et à leur appliquer, ce qui me semble plus juste, une cotisation proportionnelle au premier euro. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, ces professionnels, et particulièrement ceux qui exercent une activité saisonnière,

Il existe même des cas où la cotisation forfaitaire inciterait à ne pas travailler. Le secteur touristique est tout particulièrement touché par cette mesure, notamment les personnels appelés en renfort lors de la haute saison.

mis en place en 2015, qui a engendré une augmentation très importante de leur cotisation d'assurance vieillesse. Ce dispositif est particulièrement néfaste pour le tourisme de montagne et dissuade fortement les renforts temporaires, dont peuvent bénéficier les écoles de ski français aux périodes de pointe et dont elles ont besoin. Les moniteurs de ski occasionnels ont l'obligation d'être affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, qu'ils exercent cette activité quelques jours, voire quelques heures durant la saison ou à temps complet. Ils doivent ainsi payer 461 euros de forfait retraite, quel que soit le temps travaillé. Ce coût s'ajoute à la cotisation qu'ils payent au titre de leur première activité.

Je le maintiens,

C'est à juste titre qu'elle a provoqué beaucoup de colère dans notre pays. Dans la rue comme dans les médias, les retraités proclament partout leur malaise. Alors que les salariés vont voir leur salaire net la fin du mois d'octobre, grâce à la baisse des cotisations, eux se disent oubliés, condamnés à voir leur pouvoir d'achat s'éroder. Votée l'année dernière, la baisse de cotisations sociales pour les salariés a eu pour contrepartie une hausse de 1,7 point de CSG, qui pénalise particulièrement les retraités, et le Gouvernement y ajoute pour 2019 et 2020 une sous-indexation des pensions. Celles-ci n'augmenteront que de 0,3 % par an, quel que soit le niveau d'inflation. C'est un coup de rabot qui représente une économie pour l'État de 3 milliards d'euros en 2019. Ces nouvelles mesures s'ajoutent à de nombreux coups de canif déjà infligés ces dernières années au pouvoir d'achat des retraités : moindre revalorisation des retraites complémentaires, cotisation supplémentaire sur les pensions, décalage des dates de revalorisation La liste est longue et d'autant plus mal vécue que les retraités ne peuvent espérer compenser ces coupes par de futures augmentations de salaire. Selon Pierre Madec, économiste à l'OFCE : « À l'horizon 2020, les mesures du Gouvernement, y compris la suppression de la taxe d'habitation, vont améliorer le pouvoir d'achat d'environ 20 % des retraités. Mais pour quatre ménages de retraités sur cinq, elles aboutiront à une perte de 700 euros en moyenne, dont 600 euros du fait de la sous-revalorisation ». Conscient de la colère d'une partie grandissante des retraités, vous avez décidé de lâcher un peu de lest, mais ce n'est pas l'exclusion de 300 000 retraités qui va redonner de la justice à cette mesure. Nous proposons donc de revenir au taux de CSG antérieur à cette augmentation.

est à Mme Laurence Cohen. Dans la continuité de notre amendement précédent, nous proposons de revenir sur la fiscalisation de recettes de la sécurité sociale, en rétablissant les cotisations salariales supprimées dans le cadre du PLFSS 2018, afin d'assurer un financement solidaire et contributif des prestations sociales. En fait, les Françaises et les Français ont du mal à être convaincus qu'avec cette suppression ils voient leur salaire augmenter. Pourtant, le Gouvernement a redoublé d'efforts pour essayer de les convaincre. Mais ils

que leur pouvoir d'achat a plutôt diminué depuis la dernière élection présidentielle, et 84 % pensant que la politique du Gouvernement ne permettra pas de l'améliorer d'ici à la fin du quinquennat.

%, soit en deçà de l'inflation, et parce que les taxes sur le tabac et les carburants vont connaître au 1 janvier une nouvelle hausse. Nous proposons donc de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement de 1,7 % par la hausse de 3,4 % de la contribution sur les revenus du patrimoine et les produits de placements. Quel